pas de transition énergétique sans les collectivités territoriales. Nous avions, déposé, à une étape précédente, un certain nombre d'amendements visant à doter spécifiquement les collectivités de quelques euros par habitant pour leur permettre de faire levier

en élargissant le champ d'éligibilité des actions à celles qui présentent le meilleur effet de levier, en révisant les cibles de l'appel à projets, en créant davantage d'interaction entre les lauréats et en améliorant la cohérence de l'action de l'État. Il s'agit d'accroître le niveau d'ambition

Enfin, vous avez eu l'honnêteté de dire qu'on jouait en quelque sorte au bonneteau. Il est tout de même, me semble-t-il, assez compliqué, alors que, dans tous les territoires, on regrette de ne pas avoir assez de crédits pour l'entretien de nos routes et l'investissement, de prélever justement dans ces crédits.

de cette année. Pour la suite, c'est bien la mobilisation de tous les crédits existants- ceux de la politique industrielle et ceux du ministère de la transition écologique et solidaire -que nous souhaitons mettre en place. Nous allons accompagner les territoires d'industrie avec un volet la transition écologique. Les 124 territoires d'industrie qui ont été définis recoupent d'ailleurs largement la carte des premiers contrats de transition écologique qui ont été demandés. Ces derniers, comme l'indiquait M. le rapporteur, sont l'occasion d'une véritable contractualisation entre l'État, les établissements publics du ministère et les collectivités territoriales.

de son mandat. Cela n'est franchement pas la réponse que les Français attendent d'un débat actuel sur la transition écologique et sur la fiscalité écologique. Mme Borne nous a tenu un discours d'ancien monde,

de permettre, ce matin, à des agences de fonctionner un petit peu mieux, et cet après-midi, aux territoires qui en ont la volonté d'avoir les moyens d'assurer des missions en matière de transition écologique.

ponctuel ; elle est de savoir si l'on est capable d'accompagner un territoire dans sa globalité, avec tous les moyens disponibles des différents départements ministériels et des collectivités locales, pour que le projet de territoire soit véritablement un projet économique, écologique et

Cet amendement vise donc à concrétiser ce doublement au cours du quinquennat. Par ailleurs, le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d'importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France.

démontrer. Par rapport aux énergies renouvelables électriques, qui concentrent une très grande partie des soutiens publics, les énergies renouvelables thermiques présentent de nombreux avantages

Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement s'est engagé à porter le budget du Fonds chaleur à 315 millions d'euros en 2019, c'est bien, mais il ne prévoit pas d'augmenter le budget de l'ADEME en conséquence. Les crédits seront donc prélevés sur d'autres fonds de l'Agence, par exemple sur le Fonds déchets, alors que celui-ci finance aussi des projets de méthanisation et de valorisation du biogaz par cogénération. Où est la cohérence ? Pour sécuriser la hausse du Fonds chaleur sans obliger l'ADEME à recycler des moyens existants,

a annoncé que le Fonds chaleur, doté de 215 millions d'euros en 2018, passerait à 300 millions en 2019. Cet amendement a pour objet de concrétiser cet engagement et de transférer 100 millions d'euros, au sein du programme 181, à l'action n° 12, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin afin d'augmenter le budget du Fonds chaleur, géré par l'ADEME, opérateur de ce programme. Par ailleurs, le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d'importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France. Ce retard est notamment dû au manque d'attractivité des investissements dans ce secteur ; un projet de chaleur renouvelable sur deux finit par être abandonné parce qu'il est insuffisamment attractif. Ainsi, il est essentiel d'augmenter le montant du Fonds chaleur pour améliorer le niveau de soutien apporté à chaque projet, afin de donner aux projets de réseau de chaleur renouvelable un niveau de rentabilité suffisant. En effet, comme le souligne le Syndicat des énergies renouvelables, la chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France ; elle est pourtant aujourd'hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre.

livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030. Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d'atteindre ces objectifs.

quotidiens des transports. J'évoque spécifiquement le programme 203, « Infrastructures et services de transports », pour lequel 140 millions d'euros sont prévus, au titre de l'action Transports collectifs, pour la mise en oeuvre de ce projet.

Cette dépense, je le répète, ne nous semble pas prioritaire, alors que les besoins pour les transports du quotidien sont sous-estimés et sous-financés, ce qui conduit, en lien avec les politiques de libéralisation des transports publics, au renforcement des inégalités territoriales, qui sont au coeur

Une attention doit être spécifiquement portée aux questions d'assainissement non collectif, notamment dans les territoires ruraux. Enfin, nous considérons que des sommes supplémentaires doivent être affectées au financement du plan Biodiversité, actuellement sous-doté, particulièrement des nouvelles réserves

même si celui-ci a été réorienté, à la suite des assises de l'eau, vers le petit cycle de l'eau et les principaux investissements, l'assainissement non collectif en milieu rural reste possible, en particulier lorsqu'il s'inscrit dans une mission de service public. Encore aujourd'hui, on y consacre 10 millions à 20 millions d'euros.

non pas l'amendement, que je ne voterai pas, mais la défense du projet Charles-de-Gaulle Express, cela ne fait que renforcer ma conviction que le Gouvernement est dans l'erreur quand il veut privatiser ADP. Laissez les choses se faire selon le programme prévu, sinon vous casserez vous-même le dispositif que vous avez souhaité. Je le répète, je ne voterai pas cet amendement, car, Charles-de-Gaulle Express n'ayant pas de crédits publics en tant que tels, les crédits pourraient être retirés du budget du reste des transports collectifs, ce qui serait un désastre pour nous- ça va comme ça, c'est déjà assez difficile. Toutefois, si vous privatisez ADP, vous nous enlèverez, en Île-de-France, l'un des leviers majeurs d'intervention sur la structuration des transports publics ; et, là, franchement, je ne sais plus faire

c'est ce que le Gouvernement a annoncé en juillet dernier dans son plan Climat, et c'est ce qu'a confirmé le Président de la République mardi dernier. Pour autant, aucun dispositif d'accompagnement n'est aujourd'hui prévu, alors que les conséquences sur les entreprises, les salariés et les territoires concernés seront, bien entendu, majeures.

pour accompagner la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, à la fois pour aider les exploitants et pour aider à la reconversion des salariés et du site. Il n'y a aucune raison de traiter différemment le cas des centrales à charbon : là aussi, l'État décide d'arrêter des actifs de production bien avant leur fin de vie technique, ce qui ouvre droit à une indemnisation pour les exploitants ; là aussi, des sites industriels et des emplois disparaîtront. Il y a donc urgence à penser la reconversion industrielle de ces sites.

de créer dès maintenant une nouvelle ligne budgétaire qui permettra de financer les premières études de faisabilité des nouveaux projets d'activité économique, dès 2019. Cette ligne sera dotée de 40 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 2 millions d'euros en crédits de paiement. Il est impératif de donner de la visibilité aux industriels, aux salariés, et surtout à ces territoires. Quel est

Je veux d'abord vous rassurer, nous avons reçu les industriels. J'ai moi-même reçu le président d'EDF, la semaine dernière, et l'entretien a largement porté sur ce sujet. Le ministre d'État, François de Rugy, a reçu, avec moi, l'autre industriel, Uniper, qui est également en contact avec Bercy. Nous avons par ailleurs tenu quatre premières réunions, à Paris, avec toutes les parties prenantes. En outre, nous sommes allés à Saint-Avold et nous avons prévu de nous rendre dans chacun des sites concernés. Cet accompagnement devra faire l'objet de mesures à la fois pour les personnes concernées, qui devront être soit reclassées, soit aidées dans leur reconversion, et pour les territoires. Il n'y a pas, pour l'instant, de budget spécifique prévu. Pour la centrale de Fessenheim, je rappelle que, au-delà du protocole d'indemnisation avec EDF, le budget est pour le moment de 10 millions d'euros, en autorisations d'engagement, ce qui ne réduit pas du tout l'effort de l'État l'accompagnement du site, puisqu'un projet de territoire est en cours et appellera de nombreux investissements. Nous souhaitons faire la même chose pour les centrales de Saint-Avold, de Gardanne, de Cordemais et du Havre

industrielle et énergétique. On ne peut absolument pas rester les bras croisés et voir une entreprise comme Uniper, qui perdra d'ailleurs 56 % de sa capacité de production sur les deux centrales, disparaître de cette façon-là. Il faut que notre territoire puisse rayonner et avoir un avenir

approuvé par le préfet le 28 juin 2004. Or l'article L. 561-1 du code de l'environnement exclut le régime d'expropriation qu'il institue aux risques liés à l'érosion côtière, lesquels ne sont pas assimilables au risque de submersion marine. amendement vise donc à couvrir l'indemnisation d'immeubles situés en zone dunaire dont l'usage d'habitation est rendu impossible par le recul du trait de côte et l'érosion côtière.

cette mesure vise le cas d'immeubles à usage d'habitation dont l'accès est rendu impossible aux habitants, sans que ceux-ci soient indemnisés une procédure normale d'expropriation. À ce stade, seul l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer est concerné. N'entrant pas dans les conditions d'expropriation de l'article L. 561-1 du code précité, les propriétaires ont été tenus d'abandonner leur logement sans percevoir d'indemnités et contraints de se reloger

on les a évacués de leur logement, ils continuent à payer les charges et, aujourd'hui, ils n'ont aucune indemnisation. Il ne s'agit pas d'indemniser les membres d'autres copropriétés, il s'agit d'indemniser, dans le cadre de l'article 2, les propriétaires de cet

Nous avons tous voté à l'unanimité cette indemnité. Je ne comprendrais pas le manque de cohésion du Sénat si nous n'adoptions pas cet amendement aujourd'hui.

à bout de patience. Après les longs débats que nous avons eus, il faut agir. Agir aujourd'hui, c'est voter cet amendement, mettre le Gouvernement face à sa responsabilité, et la solidarité nationale doit jouer devant ces risques majeurs nouveaux que sont les risques environnementaux.

Je suis contre l'exonération de l'huile de palme dans les biocarburants. Néanmoins, lorsqu'il y a un moratoire et que cela peut préserver des emplois, c'est une bonne chose. Sur le CTE de Sambre-Avesnois, l'État met 12,5 millions d'euros. Pour l'instant, rien n'est prévu sur le plan financier pour le CTE de la métropole Aix-Marseille Provence. Cependant, j'aimerais connaître la nature des accompagnements que vous prévoyez pour la centrale de Gardanne : il y a le volet social,

parole est à M. Guillaume Gontard. Il s'agit encore d'un amendement de cohérence, qui a pour objet de consolider le financement des réserves naturelles nationales. Le plan Biodiversité présenté par le Gouvernement prévoit la création de cinq nouvelles réserves par an pendant quatre ans. Cette mesure n'est pas totalement financée pour l'année 2019 et nécessite un financement complémentaire de un million d'euros. Par ailleurs, pour permettre aux gestionnaires des réserves naturelles d'exercer leur mission, il convient d'augmenter le budget de un million d'euros supplémentaires. Les moyens budgétaires consacrés aux 167 réserves existantes et aux cinq nouvelles qui seront créées méritent donc d'être portés à 25,3 millions d'euros, en tenant notamment compte des subventions versées aux réserves régionales.

Il est également extrêmement curieux que les premiers subsides du plan Biodiversité ne soient pas prévus dans ce budget. L'adoption de cet amendement nous semble le minimum pour commencer à déployer les mesures de ce plan dès l'année prochaine.

pour concourir au financement du plan Biodiversité. À l'intérieur de ces 10 millions d'euros, une augmentation à hauteur de un million d'euros est fléchée pour l'extension des réserves naturelles.

300 000 euros à la protection des récifs coralliens. Je crois que nous devons aller plus loin et l'augmenter de 500 000 euros supplémentaires pour atteindre l'objectif que s'est fixé la France, à savoir protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer d'ici à 2021. Je rappelle que, à l'Assemblée nationale, cet amendement a été soutenu par les rapporteurs et que la commission du développement durable et de les récifs coralliens, joue un rôle essentiel pour promouvoir une politique active favorable à la préservation et à la gestion des écosystèmes. Elle contribue à protéger un patrimoine marin exceptionnel

La Commission nationale du débat public, ou CNDP, est l'un des acteurs qui favorisent cette information et cette association. Elle veille au respect de la participation du public dans l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national qui présentent de forts enjeux ou ont des incidences significatives sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Elle organise, vous le savez,

Par ailleurs, la Commission fait un bilan contrasté du débat public organisé de mars à juin derniers sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, justement à cause d'un manque de moyens. L'objectif est donc d'en tirer des enseignements pour le futur débat public sur le plan national

par les maîtres d'ouvrage. Dans certains cas, il s'agit de maîtres d'ouvrage privés ; dans d'autres, cela peut être le ministère lui-même. Le débat que vous avez mentionné sur les déchets radioactifs et nucléaires sera financé par la direction générale de l'énergie et du climat de ce même ministère.

Je mets aux voix l'amendement n° II-167 rectifié. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

Le scrutin est ouvert.

j'appelle en discussion les articles 75 à 76 , qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous changeons de sujet. Par cet amendement, nous souhaitons nous opposer à la baisse de la redevance nationale du permis de chasse. En effet, après avoir rencontré la Fédération nationale des chasseurs en août dernier, le Président de la République a annoncé que le Gouvernement allait diminuer de moitié le prix du permis national annuel de chasse, celui-ci celui-ci passant de 400 à 200 euros. Pour permettre cette baisse, le présent article fait passer la redevance cynégétique nationale annuelle de 197,50 euros

Dans le même temps, les redevances cynégétiques départementales sont légèrement relevées, afin de les aligner sur les redevances nationales. La principale conséquence de cette décision est financière. Le coût de cette mesure est de l'ordre de 27 millions d'euros- vous me confirmerez ce chiffre, madame la secrétaire d'État -, soit une perte de recettes de 21 millions d'euros pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. À l'heure où l'on se plaint de la disette budgétaire, comment faire l'impasse sur une telle somme ?

75 « une contribution de 5 $EUR par chasseur pour la biodiversité, associée à des cofinancements publics, pour financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité et de la restauration des habitats.

il a annoncé que le sujet serait traité dans le cadre du prochain projet de loi ordinaire relatif à la création du nouvel établissement public issu de la fusion de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et de l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité. Nous estimons que ce décalage dans le temps n'est ni souhaitable ni nécessaire. L'exposé des motifs susvisé précise bien que la baisse des redevances cynégétiques et le prélèvement sur les ressources des agences de l'eau seront compensés par cette nouvelle contribution de 5 euros. À l'heure où l'on assiste à une baisse drastique de la biodiversité, voire à son effondrement- on parle d'une sixième extinction -, ne prenons pas de retard dans les financements indispensables. Ici, la cause est belle

Cet accord prévoit notamment la réduction du prix du permis de chasse national, ce qui devrait permettre d'améliorer l'attractivité de ce permis et la mobilité des chasseurs, qui sont utiles pour maîtriser les populations de grands gibiers et réduire les dégâts

L'article 75, en ses alinéas 13 à 17, modifie les modalités de répartition des contributions des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité et à l'ONCFS. Il vient ainsi rompre avec le principe, de plus en plus détourné, selon lequel « l'eau paie l'eau ». De manière générale, la pédagogie relative aux taxes doit être plus claire si on veut le consentement.

l'eau n'ont pas à compenser la diminution des redevances cynégétiques mise en oeuvre dans le présent article. Selon certains chiffrages, le montant à compenser pourrait s'élever à 21 millions d'euros. Cette situation est d'autant plus anormale que le budget des agences de l'eau est de plus en plus contraint et qu'il paraît nécessaire aujourd'hui de le sanctuariser. Or, dans le cadre du plan 2019-2024, le plafond des recettes a été fixé fixé à 12,6 milliards d'euros sur six ans, soit une baisse de 1 milliard d'euros par rapport à la période 2013-2018. Les missions des agences de l'eau sont pourtant grandissantes et les besoins sur nos territoires impérieux, car il est nécessaire de poursuivre les travaux d'assainissement, de rénovation et de mise en conformité pour lutter contre les pollutions et préserver les ressources en eau. Partout en France, notamment dans les territoires ruraux, des communes et des collectivités territoriales ont besoin et espèrent des subventions des agences de l'eau pour pouvoir boucler financièrement leurs projets et mener à bien leurs travaux.

Les agences de l'eau, les syndicats et les associations de protection de l'environnement dénoncent cette saignée pratiquée au nom de la maîtrise des dépenses publiques. L'eau devient ainsi une simple assiette fiscale. Pourtant, compte tenu des nombreuses missions qui incombent aux agences de l'eau, il semble nécessaire de préserver le principe selon lequel « l'eau paie l'eau Cette situation est d'autant plus grave que tous les signaux de qualité de l'eau sont au rouge et que les agences de l'eau se sont déjà engagées dans des programmes ambitieux pour les six prochaines années. Les six agences de l'eau subissent aujourd'hui une telle contrainte budgétaire qu'elles ne seront plus en capacité de remplir l'intégralité de leurs missions, alors même que celles-ci se multiplient pour faire face au réchauffement climatique.

? Ce sujet reste sensible. La loi de finances pour 2018 a instauré une contribution des agences de l'eau au financement des opérateurs de la biodiversité. En contrepartie, les principales subventions pour charges de service public du programme 113 ont été supprimées, traduisant un désengagement de l'État du financement de la politique de la biodiversité. Je m'étais opposé l'an passé à ce transfert de financement injustifié aux agences de l'eau, d'autant qu'il rompait, cela a été dit, avec le principe selon lequel l'eau paie l'eau et qu'il s'éloignait également du principe du pollueur-payeur qui préside à la politique de l'eau. L'article 75 du projet de loi de finances pour 2019 ne revient pas sur cette contribution des agences de l'eau, mais il propose de nouvelles modalités de répartition de la contribution entre les agences. À ce jour, la clef de répartition de la contribution entre les agences est déterminée en fonction de la part du total des redevances.

Il est proposé que, chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartisse entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique, pondéré par l'importance relative de sa population rurale. L'adoption des amendements que nous examinons aurait pour conséquence de supprimer les nouvelles modalités de répartition de la contribution entre agences, elle n'entraînerait pas la suppression de la contribution des agences de l'eau aux opérateurs de la biodiversité, contrairement à l'intention de leurs auteurs. Cette nouvelle clé de répartition de la contribution m'apparaît

la redevance pour pollutions diffuses payée par les agriculteurs n'apporte pas de réponses concrètes à la problématique des produits phytosanitaires. L'augmentation prévue, qui consisterait à faire supporter, encore une fois, un peu plus de fiscalité

? La révision de l'assiette et des taux de la redevance pour pollutions diffuses est issue des États généraux de l'alimentation.

Mon père et mon grand-père étaient des viticulteurs bio sans le savoir, puisqu'ils n'employaient que des matières actives naturelles. Puis l'industrie chimique est arrivée, avec de nouvelles molécules

négatives de l'agriculture conventionnelle. Son impact sur la qualité des eaux, en particulier, est manifeste. Je veux réagir à l'envolée de mon collègue Daniel Gremillet

d'État, votre gouvernement a ponctionné 71 millions d'euros, en intégrant un mécanisme désormais bien connu, la fixation d'un plafond à 137 millions d'euros.

la Vendée, qui a connu la tempête Xynthia, comme nos voisins de Charente-Maritime et tout le littoral atlantique, le montant des travaux prévus pour mettre à niveau et assurer une réelle protection de nos côtes, de nos biens et de nos concitoyens s'élève à 100 millions d'euros.

toujours sur le Fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'objectif est de flécher, au sein de ce fonds, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention,

à porter la part de financement de 40 % à 60 % pour accompagner encore plus fortement les collectivités et les acteurs qui mettent en oeuvre ces travaux.

En effet, le présent compte d'affectation spéciale est alimenté par le bonus-malus, dont les recettes ont cru pour cette année de 182 millions d'euros. Nous proposons donc, et dans la continuité des annonces du Gouvernement sur un plan Vélo dans le cadre du Grand Plan d'investissement, une ligne spécifique pour l'aide à l'acquisition d'un vélo, dotée de ce supplément de recettes. Sur le fond, nous considérons que la conversion du parc automobile au tout électrique n'est pas une politique écologique suffisamment ambitieuse. En effet, si cette conversion vise à limiter les effets des gaz à effet de serre- ce n'est même pas une garantie au vu de l'explosion des ventes de gros modèles de véhicules type SUV que connaît notre pays -, elle ne remet pas en cause le nombre de véhicules individuels en circulation, et donc les problèmes de congestion automobile. L'alternative ne peut juste se situer entre la voiture et la voiture. Il faut évidemment encourager les transports collectifs, mais également les modes doux, dont le vélo à titre principal. D'autre part, le développement de la voiture électrique pose un certain nombre de questions, notamment sur les besoins en lithium. En 2040, on peut estimer que nous aurons environ 530 millions de véhicules électriques dans le monde, soit entre 150 et 200 fois plus qu'aujourd'hui. Or, actuellement, près de 35 % du lithium produit sur la planète sert d'ores et déjà à fabriquer des batteries et une telle conversion risque d'épuiser cette ressource à très court terme. Comment faire pour rendre un tel développement soutenable ? Une vraie politique écologique de transition énergétique doit donc également prendre en compte la modification de nos habitudes de mobilité. Parmi elles, il paraît judicieux de financer l'achat de vélos, électriques et non électriques. Si un vélo est un véhicule peu onéreux, le vélo électrique qui représente une solution de mobilité remarquable et les vélos particuliers du type vélo-cargo ou vélo-remorque, qui sont nécessaires pour les artisans ou les jeunes parents, sont quant à eux beaucoup plus chers et méritent de faire l'objet de cette prime. Pour ce faire, nous proposons de créer un nouveau programme, « Soutien au plan vélo », en prélevant l'équivalent de la hausse prévue pour l'année 2019, soit 182 millions d'euros,

monsieur le président. L'amendement est gagé sur des mesures qui financent à la fois la prime à la conversion et la voiture électrique. Or la prime à la conversion permet de passer à des voitures plus récentes, donc moins polluantes, quel que soit leur mode de combustion. Certes, la voiture électrique pose

spéciale « Transition énergétique », qui retrace non pas l'ensemble des dépenses que l'État affecte à la transition écologique, mais seulement certaines actions de l'État en faveur du soutien au développement d'énergies de sources renouvelables. d'affectation spéciale en 2015 a permis de donner une visibilité au Parlement sur le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité. En somme, le CAS traduit budgétairement les mécanismes de soutien : obligation d'achat d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les acheteurs et compensation pour les fournisseurs ; effacement de consommation électrique ; obligation d'achat du biométhane ... Dans Dans sa délibération du 12 juillet 2018, la Commission de régulation de l'énergie a estimé à 7 788 millions d'euros le montant prévisionnel de l'ensemble des charges de service public de l'énergie au titre de l'année 2019. 2019. Ce montant est évidemment éloigné des dépenses pour la transition écologique qui concernent tous les ministères. Ainsi, le budget du ministère de l'écologie représente environ 10 milliards d'euros, les mesures en faveur de l'efficacité énergétique du bâtiment 14 milliards d'euros sur le quinquennat, le crédit d'impôt recherche environ 6 milliards d'euros. Et il ne faut pas oublier l'ensemble des mesures d'allégement de la trésorerie décidées cette année par l'exécutif et la majorité, qui atteignent 24 milliards d'euros en baisses d'impôts

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, je commencerai mon intervention en relevant le caractère symbolique que revêt l'examen du budget de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » un dimanche après-midi Cette mission incarne le ciment de notre société. Pourtant, les annonces positives de ces derniers mois n'ont pas, me semble-t-il, été suivies d'effets : les crédits destinés au sport diminuent de 8 %, tandis que les associations sont mises sous tension du fait des réformes fiscales. Je vais concentrer mon intervention sur trois points, je dirais même trois alertes, qui méritent une attention toute particulière. La première alerte porte sur le soutien au mouvement sportif. L'année 2019 verra la mise en oeuvre d'une nouvelle gouvernance. Il s'agit d'une avancée réelle, puisque la future agence agrégera les différents acteurs et financeurs du sport. Il ne pourra toutefois s'agir d'une avancée qu'à la condition qu'on y mette les moyens nécessaires. Or, si le Président de la République s'était engagé à ce que le financement des Olympiades ne s'opère pas au détriment du sport pour tous, les chiffres révèlent une réalité différente. En 2019, puis en 2020, ce sont 20 millions d'euros d'efforts qui sont demandés au sport pour préparer l'organisation de la compétition. Il me semble difficile d'accepter que les soutiens financiers aux seules disciplines olympiques, qui sont au nombre de trente-six, se fassent au détriment des quarante-six disciplines qui Je rappelle, par ailleurs, que les dépenses du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, ont déjà subi une réduction de 63,8 millions d'euros l'an dernier du fait du transfert opéré avec le programme 219. C'est pour porter votre attention sur ce hiatus que la commission des finances a adopté l'amendement de crédits que je vous présenterai. La réponse apportée par le Gouvernement, consistant à relever de 15 millions d'euros les ressources du CNDS, n'est pas satisfaisante. Plutôt qu'un soutien effectif au sport pour tous, elle colmate les restes à payer du Centre. Ces restes à payer, dont le montant excède la centaine de millions d'euros, risquent bien de grever les moyens d'action de la future agence. La deuxième alerte porte sur le soutien aux associations. Nous le constatons tous dans nos territoires : les associations font face à de lourdes difficultés. Elles incarnent la pierre angulaire du lien social dans notre pays, mais sont pourtant minées par divers facteurs. Et les choix du Gouvernement en font partie : je pense ici à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, au profit d'un impôt à base réduite, à la réduction drastique du nombre de contrats aidés, ou encore à la diminution du concours financier des collectivités en raison de l'attrition de leurs ressources. La suppression de l'ISF, qui incitait les ménages les plus aisés à faire preuve de générosité, et un sentiment d'incertitude fiscale ont ainsi conduit ces derniers mois à une forte diminution des dons versés aux associations. Les dons pourraient chuter de 15 % en 2018, selon France générosités. La concertation engagée en novembre 2017 doit encore aboutir à des mesures concrètes, très attendues par le mouvement associatif. Peut-être pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous en dire davantage sur le calendrier La troisième alerte porte sur le service national universel, SNU. La communication a pu brouiller le message, mais soyons clairs : aucun crédit n'est prévu en 2019 pour la mise en oeuvre de celui-ci. Les crédits proposés pour le service civique correspondent à une cible de 150 000 jeunes, conforme à l'objectif fixé l'an dernier. Dès lors, évoquer une mise en oeuvre du service national universel dès 2019 s'apparente soit à une annonce erronée, soit à une insincérité budgétaire manifeste. Qu'en est-il, monsieur le secrétaire d'État ? Les obstacles sont nombreux. Ils sont juridiques, puisqu'une révision constitutionnelle est indispensable pour prévoir une phase d'engagement obligatoire. organisationnels, puisque 80 000 places d'hébergement devront être trouvées, sans que la direction de l'immobilier de l'État n'ait été sollicitée. Ils sont enfin financiers, puisque, outre un coût initial d'investissement de 1,75 milliard d'euros, le coût annuel de fonctionnement est compris entre 2,1 milliards d'euros et 4,3 milliards d'euros selon le nombre de jeunes s'engageant dans la deuxième phase. Souhaité par le Président de la République, ce service national universel soulève de nombreuses questions. Le succès du service civique dépendra des réponses qui seront apportées. Pour conclure, il me revient de vous expliquer la position de la commission des finances, qui a adopté les crédits de la mission amendés. Le soutien à la vie associative ne relève pas tant de cette mission que de dispositifs budgétaires annexes et des dépenses fiscales. Les deux autres alertes valent essentiellement pour l'avenir. En effet, la réduction des crédits du sport en 2019 est imputée par des techniques budgétaires et ne vise pas les crédits effectivement destinés au sport. L'amendement de crédits adopté par la commission des finances appelle une réponse du Gouvernement sur la trajectoire budgétaire de la mission pour les exercices à venir.

en signe de confiance dans l'action de la nouvelle équipe ministérielle et quelques semaines après l'attribution, à Lima, des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Un an après, la même commission de la culture a décidé, à l'unanimité, de donner un avis défavorable sur les crédits du sport. C'est un signal d'alarme que nous actionnons, car nous pensons que le Gouvernement n'a pas pris la mesure des enjeux et que Bercy a décidé de réduire au minimum les dotations consacrées à la pratique du sport et aux sportifs de haut niveau. Au-delà de la baisse des crédits inscrite dans le projet de loi de finances qui s'élève tout de même à 8,1 % en crédits de paiement, ce sont les incertitudes qui entourent la réforme de la gouvernance du sport qui nous conduisent Ce sont l'organisation même de la politique du sport et le rôle de ses acteurs respectifs qui vont être profondément redéfinis. Et nous sommes favorables au principe d'une évolution, allant dans le sens d'une responsabilisation des acteurs publics et privés. Mais l'annonce de la suppression du CNDS et son intégration dans la future agence nationale du sport, attendue pour 2019, posent la question du respect des engagements financiers en cours. Ainsi, les collectivités territoriales s'inquiètent pour le financement de leurs projets. Je regrette que les commissions chargées du sport dans les deux assemblées parlementaires n'aient pas été associées à cette réflexion. Nous aurions pu poser des questions sur le fonctionnement opérationnel de la nouvelle agence qui reste imprécis à ce stade, alors même qu'il nous est demandé de voter des crédits. Je pense notamment au fonctionnement des conférences régionales des financeurs et à la façon dont les collectivités territoriales et les entreprises seront associées, mais aussi à l'articulation entre l'agence et l'INSEP, Ces inquiétudes n'ont pas été apaisées, bien au contraire, par l'annonce du Gouvernement, selon laquelle l'État ne souhaiterait plus rémunérer directement quelque 1 600 conseillers techniques sportifs, les CTS. L'absence de moyens nouveaux et suffisants pour préparer les sportifs de haut niveau pour 2024 crée un doute sur les ambitions du Gouvernement.

? La commission des finances a clairement donné du corps à cette hypothèse, en constatant que 42 millions d'euros seront prélevés en 2019 et 2020 sur les crédits du sport pour financer les jeux Olympiques. Ce scénario ne serait pas acceptable, madame la ministre. C'est pourquoi nous demandons solennellement au Gouvernement de prendre la mesure des enjeux. La préparation des jeux Olympiques nécessite de produire un effort aussi physique que budgétaire, si l'on souhaite obtenir des résultats. Par ailleurs, la création de l'agence nationale du sport ne peut suffire à faire oublier le besoin d'un grand plan d'équipements sportifs à l'échelon local et la poursuite des investissements nécessaires à l'INSEP.

Mais pourquoi ne pas avoir été plus ambitieux, en déplafonnant l'ensemble des crédits extrabudgétaires qui financent le sport, en particulier le prélèvement sur les paris sportifs ? Vous n'avez sans doute pas pu, madame la ministre, peser autant que nécessaire sur ce projet de loi de finances. Nous souhaitons qu'il en soit autrement l'année prochaine. Nous ne voudrions pas que la devise des jeux de Moins vite, moins haut, moins fort madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, on peut présenter un budget en augmentation et mener une mauvaise politique C'est malheureusement ce qui caractérise les crédits consacrés au programme 163, « Jeunesse et vie associative ». Certes, je me réjouis de la poursuite du développement du service civique. En revanche, je m'inquiète de l'acharnement du Président de la République à vouloir imposer un service national universel, dont le coût paraît complètement disproportionné par rapport au bénéfice attendu. Nous en reparlerons, monsieur le secrétaire d'État. Je regrette également la stricte reconduction des autres crédits dédiés à la jeunesse et à la vie associative. Cette stagnation

par la suppression de la réserve parlementaire intervenue l'année dernière, soit 52 millions d'euros en moins pour les associations, qui n'a été compensée que partiellement à travers l'octroi de 25 millions au Fonds pour le développement de la vie associative, Je regrette donc que le Gouvernement n'ait pas augmenté cette année la contribution au FDVA. À défaut de pouvoir profiter de crédits budgétaires supplémentaires, le FDVA pourrait néanmoins voir son budget augmenter, s'il pouvait bénéficier des fonds et avoirs issus des comptes inactifs des associations en déshérence. Je proposerai un amendement sur ce sujet qui, je l'espère, recevra l'approbation du Sénat et du Gouvernement, après avoir reçu le soutien unanime de la commission de la culture. Au-delà des crédits du programme 163, la politique du Gouvernement n'est pas favorable à la vie associative et à la jeunesse. Ainsi, les avantages fiscaux et sociaux dont bénéficie le milieu associatif doivent être mis en regard de la forte baisse des crédits finançant les contrats aidés, soit une perte de 1,6 milliard d'euros de subventions indirectes pour les associations entre 2016 et 2019. Il est regrettable qu'aucune initiative ne soit prise afin d'introduire un soutien direct aux emplois associatifs au regard de leur utilité sociale, ce qui met en péril de nombreuses associations, notamment dans le domaine du sport et de la culture. Cela entraîne de graves répercussions en matière de cohésion sociale et de réponse à des besoins non couverts par les pouvoirs publics.

Hélas ! Aucune piste de réflexion n'est avancée par le Gouvernement, alors même que la fragilisation du monde associatif par la réforme des contrats aidés est accentuée par l'effet négatif des dispositions fiscales mises en oeuvre par la loi de finances pour Pourtant, qu'il s'agisse de la mise en place du service national universel, de la lutte contre la pauvreté, ou encore du développement du sport pour tous, ces exemples montrent que les associations sont censées être au coeur du dispositif gouvernemental. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez récemment fait des annonces, elles sont positives, mais elles doivent se concrétiser.

associative. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

la France a toujours été une nation donnant à la pratique physique et à la compétition sportive une place éminente au coeur de sa société. Il y a, dans notre pays, une culture active du sport qui se trouve au croisement d'importants enjeux sociétaux, sociaux et économiques. Dans ce cadre, la puissance publique est un partenaire engagé, présent aussi bien à l'échelle locale des associations sportives, qui dynamisent nos territoires et constituent un fort levier de cohésion sociale, qu'à l'échelon international du sport de haut niveau, garant du rayonnement et de l'influence de la France. De grands chantiers se trouvent aujourd'hui engagés, et ils représentent de fortes opportunités pour le constant développement de la culture et de la pratique sportives. Les jeux Olympiques de 2024 constituent bien sûr un rendez-vous majeur. L'événement donnera à notre pays et à sa capitale une visibilité considérable. Nous connaissons tous les enjeux économiques et d'influence qui sont liés à l'organisation des jeux Olympiques, mais il convient d'aller plus loin et de souligner à quel point cet événement sportif constitue un catalyseur en matière, par exemple, de développement des infrastructures et des transports. Les jeux Olympiques créent du lien, de toutes les manières possibles. La réussite de ces jeux Olympiques et Paralympiques ne passera pas seulement par le nombre de médailles récoltées. L'engouement qu'ils susciteront dans notre pays est une opportunité, dont il faut se saisir, pour amener vers la pratique sportive ceux qui en sont, ou s'en sont, éloignés. Je rappelle que l'ambition a été affirmée jusqu'au sommet de l'État de porter le nombre de pratiquants à 3 millions d'ici à 2022.

Je ne doute pas que vous aurez l'occasion d'éclairer la chambre haute sur les missions et la forme de cette agence. J'ajoute simplement que, si le CNDS avait quelques défauts, dont celui d'avoir accumulé quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros de factures impayées, il avait aussi le mérite d'avoir fortement soutenu la pratique sportive, notamment dans nos territoires. Je formule ainsi le voeu, madame la ministre, que ce lien étroit avec les territoires ne soit pas rompu avec la création de l'agence et que son action s'inscrive, au moins sur ce plan, dans la droite ligne d'une coopération renforcée avec les élus et les associations. les associations. Une ambition commune s'affirme à travers ces chantiers : démocratiser la pratique sportive et la rendre non seulement plus accessible, mais aussi plus évidente. Et nous pouvons nous réjouir de la double volonté de renforcer le nombre de licenciés dans les clubs, celles et ceux qui constituent le terreau fertile sur lequel éclosent les champions qui font rayonner le France, et d'inciter un nombre croissant de personnes à faire du sport, un indispensable facteur de santé, de bien-être et de plaisir.

médaillés olympiques, et non des moindres, se sont adressés au Président de la République et aux élus de la Nation, s'inquiétant d'une possible remise en cause des moyens alloués aux fédérations et d'une baisse du budget du ministère. Si nous ne pouvons que souscrire à leur volonté de voir la France conserver sa place dans le concert des grandes nations sportives, voire de l'améliorer, si nous devons entendre ces inquiétudes, il faut aussi examiner les moyens alloués à travers le prisme de la réforme en profondeur de notre politique sportive, sur laquelle je m'exprimais à l'instant. La question qui guide la majorité et le Gouvernement depuis le début de ce quinquennat est en effet de savoir non pas s'il faut dépenser plus, mais comment dépenser mieux. bien, déjà, les critiques de nos collègues qui nous accusent de mettre à mal le modèle sportif français à la lumière de cette diminution constatée du montant du budget des sports. Cette diminution, cependant, j'oserai

Nous devons par ailleurs garder à l'esprit la disparition en début d'année prochaine du CNDS, remplacé avant l'automne par l'agence nationale du sport, l'ANS. Chacun imagine bien que le CNDS n'engagera pas d'argent en début d'année, sachant sa disparition proche, et alors que l'ANS sera à même de reprendre cette activité mi-2019, selon toute vraisemblance. Les moyens de cette nouvelle agence sont non seulement préservés, mais également augmentés, puisque le Gouvernement et Mme la ministre nous proposent d'augmenter de 55 millions d'euros les fonds alloués, d'une part, à la haute performance, et, d'autre part, au développement des pratiques. Ce sont 25 millions d'euros d'un côté, 30 millions d'euros de l'autre, au bénéfice de la nouvelle agence nationale du sport, qui sera ainsi portée sur les fonts baptismaux sous les meilleurs auspices. D'une manière générale, avec ce budget des sports, il convient de souligner la volonté du ministère de réorienter son action vers les pratiquants en général, et de mieux répartir les moyens entre le sport professionnel et le sport amateur. Ce budget manie l'ambition « en même temps » de donner aux sportifs les moyens de s'épanouir, à tout niveau, dans leur discipline, et d'engager, avec toute la prudence requise lorsque l'on gère l'argent public, les fonds nécessaires pour leur donner cette possibilité. Aucun moyen n'est donc ôté au milieu sportif, comme on a pu l'entendre dire par ailleurs, ou comme certains grands sportifs ont pu s'en inquiéter. Plus de projets pourront être menés en 2019, et, par effet de levier, nous savons bien que les collectivités locales, d'ailleurs souvent subventionnées par l'État, alimentent largement les budgets des associations, directement sur le terrain. Je crois donc pouvoir affirmer, avec l'ensemble de mes collègues du groupe La République en Marche, que le budget que nous propose d'adopter le Gouvernement est à la hauteur de toutes nos ambitions et qu'il servira les intérêts de toutes celles et de tous ceux qui contribuent à diffuser toujours davantage la culture sportive au coeur de notre société.

C'est tout à fait contradictoire avec l'ambition affichée d'aller vers 3 millions de sportifs supplémentaires, et cela risque de donner un goût amer aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, comme aux autres grandes compétitions que la France accueillera dans les prochaines années.

inquiètent de nombreux acteurs, jusqu'à provoquer une réaction sans précédent du mouvement sportif, tant de la part des professionnels que des bénévoles. L'augmentation des crédits destinés au sport professionnel et de haut niveau ne masque pas les ponctions, à hauteur de 40 millions d'euros, sur le sport amateur. Derrière ces chiffres, je l'affirme, il y a la volonté de mettre fin au modèle français du sport populaire, amateur, représenté notamment par 3,5 millions de bénévoles engagés dans leurs clubs locaux, dans nos villes, nos quartiers comme nos villages, au profit d'un modèle d'inspiration britannique, un modèle centré sur la performance, le haut niveau, où la salle de sport offre un service payant à ses clients, en lieu et place d'une licence dans un club ou une association. Ce modèle démontre outre-Manche son incohérence et son inefficacité. En effet, assécher le sport de masse, c'est, à terme, se priver de la performance et du plus haut niveau. C'est pourtant ce chemin que nous risquons d'emprunter, l'État n'entendant plus assumer sa mission de définition d'une politique sportive ni assurer le service public déclinant

Ces CTS jouent pourtant un rôle essentiel dans la formation des éducateurs sportifs, la détection des jeunes talents et les plans locaux de développement du sport. Je mets le terme « transfert » entre guillemets, car nous avons bien noté que, face au mécontentement, le Gouvernement a indiqué que ces conseillers seraient non pas supprimés, mais réorientés. imaginer que les fédérations pourront les accueillir et les financer est tout simplement irresponsable, tout particulièrement dans un contexte où, cette année encore- faut-il le rappeler ? -, les associations sportives souffriront de la disparition des contrats aidés.

À affaiblir constamment le sport public, c'est son versant privé que l'on favorise, comme je l'ai déjà dit. Il vaudrait mieux libérer le sport de l'argent plutôt que d'y faire entrer davantage d'intérêts mercantiles. Cette évolution est renforcée par la diminution des moyens des collectivités territoriales. Elles investissent plus de 12 milliards d'euros par an dans le sport, mais les premiers effets des baisses de dotations qu'elles subissent se font sentir, puisqu'un quart d'entre elles ont déjà diminué leurs subventions au sport. Au bout de la chaîne, les clubs, pour subsister, n'auront d'autre choix que d'augmenter le prix des licences. C'est évidemment impensable, sauf à vraiment refuser d'entendre le cri de colère de la France sur le pouvoir d'achat. Quant aux 15 millions d'euros accordés à la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive sur les territoires carencés, axés notamment sur la natation, ce montant est si faible pour des enjeux si importants que cela n'est tout simplement pas sérieux. Enfin, une des portes d'entrée dans la pratique sportive, c'est l'éducation physique et sportive, l'EPS. Là non plus, les perspectives ne sont pas brillantes. Toujours pas d'épreuve finale au baccalauréat, et la réforme du lycée amène à faire de l'EPS la seule discipline du bloc obligatoire à ne pas avoir de spécialisation. Je terminerai, trop brièvement malheureusement, en évoquant les crédits de la jeunesse et de la vie associative. L'équation est une nouvelle fois simple : l'intervention de l'État, concentrée sur le service civique, ne vient même pas compenser la baisse des dons induite par la suppression d'une part importante de l'ISF, la diminution considérable des emplois aidés et la multiplication des missions que l'État confie aux associations, la ligne budgétaire consacrée au développement de la vie associative diminuant même d'un million d'euros. Vous ne serez donc pas surpris que le groupe CRCE vote contre ce budget. La parole Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous évoquons ce jour les crédits alloués à la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances. Sur le volet sportif, l'an passé, nous déplorions un recul des moyens d'environ 7 %. L'essentiel de cette baisse a touché la part territoriale du CNDS. Le budget qui nous est soumis pour 2019 s'inscrit dans la même tendance au repli. L'effort consacré à la pratique sportive dans nos territoires semble une nouvelle fois pâtir des moyens mobilisés pour accueillir les jeux de la XXXIII Olympiade en Île-de-France et à Marseille. C'est un signal particulièrement inquiétant, au moment où la désaffection populaire pour ce type de manifestation est toujours plus significative. Pour mémoire, après quatre référendums perdus par des comités d'organisation, seule la ville de Milan est aujourd'hui un candidat certain pour accueillir les jeux Olympiques d'hiver en 2026. Comment prétendre faire des jeux Olympiques en France un succès populaire si la concrétisation de ceux-ci est perçue comme faite au détriment du sport pour tous, que les valeurs olympiques sont pourtant censées aussi promouvoir ? Le groupe du RDSE soutient donc pleinement la proposition réitérée par notre collègue rapporteur pour avis, Jean-Jacques Lozach, d'élaborer une loi de programmation budgétaire dédiée à cet événement et à la Coupe du monde de rugby, qui le précédera d'un an. Il est nécessaire de sanctuariser les moyens alloués à ces manifestations, en isolant notamment les crédits alimentant la SOLIDEO, pour ne pas risquer de compromettre l'image de ces jeux, qui ont avant tout vocation à valoriser la pratique sportive dans notre pays.

Le second point d'inquiétude des élus du groupe du RDSE porte sur la réforme de la gouvernance du sport à venir. Nous sommes convaincus de l'utilité de la démarche, alors que la pratique sportive, amateur comme professionnelle, a connu de profondes mutations ces dernières années. Toutefois, cette réforme ne doit pas conduire l'État à se désengager progressivement du financement et de la gouvernance du mouvement sportif., les dépenses supportées par le programme 219 et le CNDS devront donc être maintenues au sein de la future structure. Nous nous interrogeons, en outre, sur l'avenir même du ministère des sports après 2020, lorsque la nouvelle agence sera pleinement opérationnelle. Ce désengagement devrait également se traduire par la suppression de 1 600 conseillers techniques sportifs à l'horizon 2022, ce qui représente plus de la moitié des agents du ministère. Compte tenu de l'ampleur de la réforme envisagée, nous souhaiterions disposer enfin d'informations plus détaillées, tout particulièrement sur l'association des collectivités territoriales, des fédérations et des entreprises au sein de la future agence. Sur le volet jeunesse et vie associative, nous constatons la montée en puissance du service civique, qui sera en mesure d'accueillir 140 000 volontaires l'an prochain. Nous continuons d'apporter notre soutien à ce dispositif créé en 2010. Nous demeurons en revanche beaucoup plus réservés sur la perspective de concrétiser l'engagement du Président de la République sur la mise en oeuvre d'un service national universel, compte tenu du coût très important du déploiement de celui-ci. Concernant la vie associative, force est de constater, en dépit de multiples mises en garde, que le Fonds pour le développement de la vie associative, qui ne fait pas l'objet d'une revalorisation dans ce projet de loi de finances, est très loin de pallier la disparition de la dotation d'action parlementaire. Contrairement à ce qui avait été annoncé à la représentation nationale, les montants alloués précédemment à la réserve parlementaire n'ont pas été reconduits sous d'autres formes. Dans le même temps, la forte baisse des crédits relatifs aux contrats aidés se poursuit, alors que 40 % d'entre eux bénéficient aussi aux associations. Comme l'a très justement rappelé notre rapporteur, cet assèchement équivaut à la suppression de 1,5 milliard d'euros de subventions indirectes.

de manière bénévole ou quasi bénévole, de poursuivre leur engagement faute de moyens suffisamment adaptés. Ne sous-estimons pas le rôle crucial joué par ces derniers dans la cohésion nationale. Mes chers collègues, ce projet de budget comporte des points positifs. Toutefois, les motifs d'inquiétude qu'il suscite sont trop prégnants pour ne pas être mis en avant. J'attire l'attention des membres du Gouvernement sur l'unanimité qui a prévalu à la commission de la culture de la Haute Assemblée au moment d'émettre un avis défavorable sur l'adoption des crédits de cette mission.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est au nom de mon collègue Claude Kern, qui a dû s'absenter, que je m'exprime devant vous. La mission « Sport, jeunesse et vie associative » voit cette année ses crédits augmenter de près de 4,1 %, soit plus de 39,7 millions d'euros supplémentaires. Si nous saluons cette hausse, la diversité des thématiques réunies ici impose de regarder davantage dans le détail. Ainsi, le programme dédié au sport connaît un recul de 8,1 %, pour atteindre 319,2 millions d'euros. Madame la ministre, vous aviez défendu, lors de vos auditions, un budget préservé pour les sports, justifiant la baisse des crédits de votre ministère par des ajustements techniques. Cependant, cette baisse s'annonce lourde de conséquences pour le monde sportif français. En effet, la diminution du budget dédié à la promotion du sport pour tous de 44,9 44,9 % est particulièrement alarmante. Je n'ai pas besoin de vous convaincre du rôle social extrêmement important que les clubs de proximité jouent dans nos villages et dans nos villes, dans nos quartiers et dans nos territoires, en particulier les plus délaissés. Ils constituent des lieux de sociabilité pour les jeunes, comme pour leurs familles, et participent de l'éducation de nos enfants à travers la promotion des valeurs éducatives, sociétales

haut niveau français, alors que se profilent les jeux de Tokyo en 2020, puis, surtout, de Paris en 2024. Il s'agit de préparer nos sportifs de haut niveau à l'excellence, si nous voulons en faire de vrais champions. Or tout champion, quelle que soit sa pratique, a nécessairement commencé un jour au club de son village ou de son quartier, club qui l'a ensuite accompagné tout au long de son parcours. L'augmentation du budget dédié au sport de haut niveau, de 4,6 %, n'est donc à ce titre qu'une demi-satisfaction, tant elle est altérée par l'opposition créée entre deux pratiques qui sont pourtant complémentaires. Au-delà du strict examen budgétaire, de nombreuses questions soulevées dans le cadre de cette mission restent sans réponse. Ainsi, quel sera l'effet de l'intégration du CNDS au sein de la future agence nationale du sport sur les financements des clubs et associations ? Cette agence devrait reprendre en effet le budget du CNDS, bras financier du ministère des sports chargé d'en répartir les financements, soit 130 millions d'euros. de la répartition des aides à l'avenir ? Les 15 millions d'euros supplémentaires votés en première partie du PLF vont-ils réellement servir au sport pour tous, comme cela a été évoqué en commission à l'Assemblée nationale, ou plutôt à payer les restes à charge du CNDS, comme cela a été soutenu en séance publique, toujours à l'Assemblée nationale ? De même, les inquiétudes sur le devenir des 1 600 conseillers techniques sportifs n'ont pas encore trouvé de raison de s'apaiser. Je veux parler du transfert de ces CTS vers les fédérations et les collectivités, alors que la grande majorité n'aura pas les moyens de se payer un cadre d'État, solution par ailleurs inacceptable. Ces agents jouent pourtant un rôle extrêmement important dans le monde sportif, notamment dans la démocratisation du sport, la formation des cadres sportifs et la détection de nouveaux talents, qui porteront haut les couleurs de la France. Leur disparition risque fort de rajouter à la fracture entre sport de haut niveau et sport et sport de proximité. Nous nous acheminons donc vers une politique à deux vitesses, en contradiction avec le principe d'un service public à destination du plus grand nombre. Le sport n'est pas le seul domaine concerné par cette mission. La jeunesse et la vie associative voient ainsi leur budget, rattaché au ministère de l'éducation nationale, augmenter de 8,9 %, pour atteindre 614 millions d'euros. À ce titre, nous saluons l'effort significatif porté sur le service civique. Cependant, la diminution des crédits dédiés au développement de la vie associative, qui étaient déjà faibles, doit être mentionnée. Les associations, nous le savons, sont essentielles à notre cohésion nationale, mais force est de constater que, si on leur demande beaucoup, on leur donne peu. J'en profite pour saluer l'action et le dévouement des nombreux bénévoles au service de notre jeunesse, notamment. La suppression de la réserve parlementaire vient encore aggraver cette situation, et ce d'autant plus que le FDVA, censé la remplacer, ne dispose que de la moitié de ses moyens. De plus, l'attribution des aides manque de transparence. Une fois encore, la mission que nous examinons aujourd'hui, en particulier son volet sport, sert de variable d'ajustement budgétaire. Cela est difficilement supportable, dans la mesure où le budget dédié au sport ne représente que 0,13 % du PIB, ce qui est objectivement très peu au regard des enjeux que représentent l'organisation des jeux Olympiques de 2024 ou, plus généralement, le rôle du sport dans la société, notamment Je le dis sans ambages, madame la ministre, le Gouvernement n'a pas choisi la bonne méthode. Alors même que la France ambitionne de ramener quatre-vingts médailles des prochains jeux Olympiques de 2024 et vise une augmentation sans précédent du nombre de licenciés, il faut se donner les moyens de nager dans dans le grand bain, si vous me permettez de reprendre cette expression. Des efforts doivent donc être entrepris, et ce dès maintenant. Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste, que je représente, ne votera pas le budget de cette mission en l'état, car les moyens présentés ne sont pas à la hauteur des ambitions.

messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » connaissent une hausse de 22,3 % en autorisations d'engagement et de 4,1 % en crédits de paiement par rapport à l'année dernière. La hausse globale de l'enveloppe budgétaire masque des évolutions hétérogènes au sein de la mission. Si le financement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et les dépenses du service civique captent l'essentiel des crédits, le programme sport, hors jeux Olympiques, connaît une attrition de plus de 8

et de bonne gestion financière, il ne faudrait pas que nous en arrivions à réduire certaines mesures visant à promouvoir les pratiques sportives ou à ne pas accompagner les petits clubs sportifs. Nous suivrons avec attention la mise en place de l'agence nationale du sport au 1 mars 2019. Cette structure remplacera le Centre national pour le développement du sport. Ces objectifs doivent bien être complémentaires le travail mené pour les jeux Olympiques de Paris en 2024 doit se faire en parallèle avec la promotion de la pratique d'activités sportives. L'objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici à 2022 est ambitieux, mais doit être atteint. Cette agence doit notamment être pourvue des moyens financiers nécessaires, notamment pour ce qui concerne le sport pour tous et les nouvelles mesures en faveur de la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive sur les territoires carencés. Nous resterons aussi vigilants sur l'avenir des 1 600 conseillers techniques sportifs, pour lesquels les annonces du Gouvernement ont ont suscité des inquiétudes dans le milieu sportif. Nous soulignons également qu'il ne faut pas négliger le soutien aux petites associations sportives- je suis issu du milieu rural et je les connais particulièrement bien -, qui doivent qui doivent faire face à un contexte difficile, alors qu'elles assurent le maillage territorial de nombreuses pratiques sportives. La conciliation entre l'organisation des jeux Olympiques et la maîtrise des comptes publics ne doit pas s'opérer au détriment des associations de nos territoires. Les jeux de 2024, qui seront sans conteste un grand événement pour la France et ses territoires, ne seront une réussite qu'avec la participation active du tissu sportif de terrain. la France est riche, en plus de son tissu sportif, de plus d'un million d'associations, animées par 13 millions de bénévoles passionnés et 80 000 jeunes en service civique. Les salariés du secteur représentent 9,7 % des salariés du privé. le tissu associatif pâtit de la suppression de la réserve parlementaire et de la baisse du nombre de contrats aidés, qui ont dégradé les conditions de fonctionnement et de financement de bon nombre d'associations locales. La France ne peut se concevoir sans l'engagement de ces citoyens, qui ne comptent pas leurs heures ni dans leur portefeuille pour donner du temps, de la compétence et faire preuve de générosité. collègues, le tissu associatif est le ciment de la République, le dernier rempart contre l'isolement, le populisme et la montée des égoïsmes. Si l'État ne peut être partout, il doit cependant prendre ses responsabilités pour valoriser l'action de ceux qui agissent là où il ne peut lui-même aller, au coeur du terrain, au plus près des besoins et des initiatives. La majoration de 25 millions d'euros de la dotation du Fonds pour le développement de la vie associative permettra de compenser, partiellement seulement, la suppression de la réserve parlementaire, mais cela reste insuffisant pour pallier la diminution des contrats aidés et la fragilisation des ressources des plus petites associations. J'ai été longtemps élu local, et j'ai

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici réunis aujourd'hui afin de débattre du budget de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Mon intervention se concentrera sur le budget des sports pour 2019. bien consciente, l'ambiance actuelle dans le milieu sportif est à l'inquiétude et au désarroi. Le mouvement sportif s'interroge sur son organisation ; les bénévoles sont désemparés et les responsables locaux arrivent difficilement à gérer les demandes quotidiennes toujours plus nombreuses et toujours plus contraintes. Votre ministère a également du retard sur de nombreux dossiers. L'Agence française de lutte contre le dopage ne connaît toujours pas votre arbitrage sur son futur site, alors qu'il s'agit là d'un outil de rayonnement français très fort. Le préfigurateur de l'ANS n'est toujours pas nommé, alors que celle-ci est censée être à pied d'oeuvre au 1 mars. La stratégie relative au sport de haut niveau demeure floue. Quant à la politique du sport pour tous, rien n'est défini en matière d'objectifs et de moyens. Le statut des CTS et leur évolution ne sont toujours pas réglés, et le sport scolaire attend une réponse à une demande de moyens supplémentaires, afin de mieux fonctionner pour s'inscrire dans la dynamique des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il y a ainsi de nombreux exemples. Sans vouloir opposer les domaines, je constate que le sport est le grand perdant des politiques nationales, et les signaux négatifs s'amoncellent pour un pays qui devrait être totalement mobilisé pour préparer au mieux les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 suppression de l'option sport au baccalauréat ; suppression des emplois aidés ; suppression de la réserve parlementaire ; baisse des moyens des collectivités, qui sont les premiers financeurs du sport. Et le budget que vous nous présentez pour 2019 est une nouvelle fois en diminution. Certes, vous avez comblé les trous à l'Assemblée nationale, mais il manque toujours 15 millions d'euros pour atteindre le niveau de 2018.

vous nous soumettez aujourd'hui en dernière minute un amendement qui a pour objet de réduire de près de 2 millions d'euros le budget du sport, ce qui conduira à une baisse de 17 millions d'euros par rapport à 2018.

Une des demandes légitimes du mouvement sportif est de déplafonner les taxes affectées au sport. Que le sport finance le sport ! Il est en effet totalement anormal que ces taxes créées pour le financement du sport soient finalement fléchées en grande partie pour combler les erreurs budgétaires du Gouvernement. Chaque année, leur montant augmente et, chaque année, la part reversée au sport diminue. Je rappelle aussi le détournement sur le dos de Paris 2024 du prélèvement complémentaire de 0,3 % sur les mises sur les jeux. Ce prélèvement,

par le fait du prince, à la suite d'un coup de téléphone, la Fondation du patrimoine se voit reverser toutes les taxes issues de son nouveau jeu de grattage. Tant mieux pour elle, mais ce qui est possible pour le patrimoine devrait l'être pour le sport. Autre exemple, madame la ministre, vous avez évoqué devant notre commission un plan « piscine et anti-noyades ». Nous y sommes favorables, mais soyons honnêtes, le budget que vous présentez ne permettra pas de soutenir la réhabilitation,

C'est l'organisation même de la politique du sport et le rôle de ses acteurs respectifs qui vont être profondément redéfinis à la suite de la consultation menée depuis janvier 2018 sur la rénovation du modèle sportif français. Différentes réflexions ont, par ailleurs, été conduites ces derniers mois. Je pense notamment au groupe de travail de Claude Onesta « Performance 2024 ». La création de la future agence nationale du sport, qui sera effective au 1 mars 2019, suscite aujourd'hui des espoirs, mais également des craintes, certains experts mettant en évidence le risque de privatisation de la politique en faveur du sport et le fait que l'État pourrait renoncer à exercer pleinement une mission essentielle qui lui incombe. Sans reprendre nécessairement cette analyse à notre compte, nous considérons que les incertitudes qui demeurent écornent, à ce stade, le droit d'information du Parlement. Ces inquiétudes concernent également l'annonce du Gouvernement selon laquelle l'État ne souhaite plus rémunérer directement quelque 1 600 CTS. Même si cette évolution n'est pas prévue dans le présent projet de loi de finances, la réaction a été vive dans le mouvement sportif, comme en témoigne la lettre ouverte aux élus, signée par près de 400 sportifs de haut niveau. La mobilisation a été d'autant plus forte que la réduction drastique des contrats aidés et la suppression en région de nombreux emplois associatifs ont aussi fragilisé et vont encore plus fragiliser dans l'avenir le maillage territorial des clubs.

Faute de pouvoir disposer de cet outil qui sanctuariserait les moyens nécessaires à l'organisation de ces grands événements, le risque est réel que la baisse des crédits du programme 219, suite d'ajustements, ne soit perçue comme un transfert de crédits vers le programme 350, ce qui pourrait nuire à ce grand événement populaire que doivent être les jeux Olympiques et Paralympiques. En matière d'équipements, la nécessaire rénovation du Stade de France, futur stade olympique en 2024, avait été évaluée dans un premier temps à 50 millions d'euros dans le protocole financier des Jeux

Pour autant, nous avons bien conscience de la nécessité d'actualiser, de moderniser le modèle sportif français en intégrant le phénomène de mondialisation, l'hyper-médiatisation, la diplomatie sportive. Il est urgent d'avancer afin de répondre à l'explosion du sport-business dans certaines disciplines, à la montée en puissance des collectivités territoriales, à la nécessité de densifier le sport-entreprise en associant le monde économique, à l'autonomie attendue du mouvement sportif.

La mise en oeuvre d'une stratégie ambitieuse en matière de sport-santé demeure un enjeu majeur de santé publique et, à mes yeux, la porte d'entrée la plus pertinente pour accroître le nombre de pratiquants. Or une telle orientation ne se dégage pas clairement du budget. Plus généralement, le sport doit contribuer à l'activité économique, à l'emploi, à une société plus inclusive, ce qui implique de moderniser la mission de service public déléguée par l'État. Dans le nouveau schéma d'organisation, il est prévu que les services du ministère recentrent leur action sur les missions de stratégie, de régulation, de réglementation et de contrôle, notamment éthique.

La réussite de la mutation en cours se mesurera en particulier à l'aune des résultats des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous devons être à la hauteur de l'enjeu tant pour l'organisation que pour le nombre de médailles. Nous avons une double obligation de résultat. J'observe que le Gouvernement a souhaité commencer par réformer l'organisation du sport français. Je souhaite qu'il s'attelle demain aux moyens, afin de ne pas faire l'impasse sur les jeux Olympiques d'été de 2020 et les jeux Olympiques d'hiver de 2022, sans oublier les autres rendez-vous internationaux avant 2024. Le 13 septembre 2017, la France obtenait l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, soulevant un grand enthousiasme dans le pays. La préparation de ces jeux nécessite de construire d'ici à 2024 un « héritage olympique », qui fait aujourd'hui consensus. la ministre, les ambitions de votre prédécesseur- quatre-vingts médailles pour la France et un accroissement de trois millions du nombre de pratiquants. Pour atteindre ces objectifs, des moyens financiers et humains doivent être à la hauteur des enjeux. depuis le 13 septembre 2017, après un budget des sports pour 2018 en baisse, le Gouvernement nous propose de nouveau un budget en diminution. Par ailleurs, nous comprenons difficilement pourquoi les 481 millions d'euros des crédits du budget pour 2018 n'ont pas été intégralement consommés.

Concernant le programme « Jeunesse et vie associative » de la mission, il nous paraît regrettable qu'aucune initiative ne soit prise, afin d'introduire un soutien direct aux emplois associatifs au regard de leur utilité sociale, ce qui met en péril de nombreuses associations, notamment dans le domaine du sport et de la culture, et entraîne de graves répercussions en matière de cohésion sociale et de réponse à des besoins non couverts par les pouvoirs publics. Plusieurs pistes sont envisageables : créer un fonds qui s'inspirerait du FONJEP et qui permettrait de financer du personnel associatif auprès des associations créer une ligne budgétaire spécifique au sein du fonds d'inclusion dans l'emploi, permettant le financement de 38 000 emplois utiles socialement, afin de soutenir la professionnalisation des projets associatifs, tout particulièrement dans les petites et moyennes associations. Je vous rappelle que la fragilisation du monde associatif avec la réforme des contrats aidés est accentuée par l'effet négatif des dispositions fiscales mises en oeuvre par la loi de finances pour 2018. Pourtant, qu'il s'agisse de la mise en place du service national universel, de la lutte contre la pauvreté, ou encore du développement du sport pour tous, pour ne prendre que ces trois exemples, les associations sont censées être au coeur du dispositif gouvernemental. Il est donc urgent que le Gouvernement donne un signal positif en direction des associations et les soutienne dans le financement des missions d'intérêt général qu'elles remplissent.

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2019 s'inscrit dans la préparation des grandes échéances sportives organisées par notre pays ces prochaines années Coupe du monde féminine de football en 2019, Coupe du monde de rugby en 2023, Mondiaux de ski à Courchevel-Méribel en 2023, mais, surtout, jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Bien entendu, le spectre d'un financement des Olympiades 2024 au détriment du mouvement sportif plane déjà au-dessus de nos têtes. Pour l'éloigner ou tenter de le masquer, on nous annonce, à grand renfort de communication, des crédits en hausse, conformément à la trajectoire du budget triennal. triennal. Au-delà des effets d'annonce, qui ne trompent plus personne, et des manipulations de chiffres, dans lesquels le Gouvernement est passé maître, cette augmentation est, en vérité, uniquement le fait de deux facteurs principaux : les dépenses du service civique inscrites au sein du programme 163 et et les besoins de financement au titre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous y voilà ! La comparaison entre, d'une part, la trajectoire budgétaire pour les années 2018 à 2022 précédant l'attribution des Olympiades de 2024 à la France et la trajectoire actualisée pour tenir compte de l'organisation de la compétition, et, d'autre part, les besoins de financement constatés sur le programme 350, « Jeux olympiques et paralympiques 2024 2024 », fait apparaître un écart non compensé de plus de 20 millions d'euros, chaque année, pour 2019 et 2020. La réalité brutale, c'est que les les crédits de paiement du programme 219, « Sport » diminuent clairement de plus de 8 % par rapport à 2018. C'est une honte ! À l'heure où l'on tague l'Arc de Triomphe, il n'est pas un jour, pas une minute sans que l'on ait besoin, de façon urgente, de consolider trois piliers indispensables au bon fonctionnement de notre société, malheureusement déstabilisés aujourd'hui : la santé, l'éducation, l'intégration. Quel domaine, mieux que le sport, permet de répondre grâce à un seul et même vecteur à ce besoin urgentissime ? Madame la ministre, quel domaine mieux que le sport est capable de redonner sens au mot si beau et si profond qu'est le mot « nation », le mot « nation », que des apprentis sorciers vident de son sens premier pour mieux racoler honteusement ? Les fonctions éducatives et sociales portées par le mouvement sportif dans nos territoires, en lien avec un encadrement de qualité, contribuent avec force et vigueur aux missions d'intérêt général et de service public. Le sport mérite mieux que les coups de rabot dévastateurs portés par Bercy chaque année ! Si la France affiche des objectifs ambitieux en matière sportive et si notre pays veut enfin devenir la grande nation sportive dont nous rêvons tous, il faut changer de braquet Autre victime collatérale des restrictions budgétaires, les aides en faveur des territoires. Disons-le honnêtement, ce budget pour 2019 ne permettra pas de répondre aux besoins en équipements de nombreuses communes. La forte baisse de la part territoriale du CNDS en 2018, c'est moins 50 % de subventions à la base du sport sur l'ensemble du territoire. Depuis dix-huit mois, votre politique remet en cause, mesure après mesure, cet idéal sportif qui devrait nous rassembler. Fragiliser les associations sportives qui font un travail exceptionnel aux côtés des fédérations nationales, c'est briser la chaîne qui nous rassemble autour de l'effort, de la solidarité et de l'ambition. Le FDVA n'est crédité que de 25 millions d'euros au titre de sa nouvelle mission de financement des associations et ne saurait compenser la suppression de la réserve parlementaire. La diminution des contrats aidés, dont un tiers concerne le secteur associatif, a elle aussi frappé de plein fouet le monde sportif, et ce alors même que les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 suscitent un élan sans précédent chez les bénévoles

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter cet après-midi, dans le cadre de l'examen de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », le budget pour 2019 du programme 219, « Sport » et du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 d'abord d'un budget préservé, dont je veux souligner la cohérence ; un budget cohérent, car il s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de respecter ses engagements budgétaires et de se positionner dans une action efficiente. aussi un budget fidèle, fidèle aux deux grands objectifs que nous avons définis avec le Président de la République et le Premier ministre. Le premier objectif est de réussir les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous devons livrer des infrastructures dans les délais et dans le cadre de coûts raisonnables. Cette volonté de réussite se traduit actuellement par les crédits affectés au programme 350.

2018. La réussite des Jeux devra aussi et surtout être évaluée à la lumière de notre performance sportive et sociale. Vous le savez, après Rio, nous avons fait le constat que notre système de détection et d'organisation du sport de haut niveau était performant. Toutefois, nous devons améliorer la haute performance, la dernière marche vers la réussite. Cette haute performance se fabrique par l'athlète et son entraîneur. Ce sont eux qui ne sont pas, aujourd'hui, suffisamment aidés. La cellule « athlète-entraîneur » doit être l'objet de toute notre attention ; ce duo doit être accompagné de manière optimale, tant dans son objectif de médailles que dans sa reconversion. Les Jeux réussis, c'est aussi l'assurance de toutes et de tous de profiter de leurs retombées positives dans notre pays. Je souhaite, pour cela, passer du « ministère de ceux qui font le sport » au « ministère de ceux qui font du sport ». Les fédérations seront, bien entendu, au coeur du dispositif, mais elles ne seront pas les seules. Les acteurs non affiliés au système fédéral devront également mieux être pris en compte, tout comme le développement territorial du sport. Nous entendons d'abord mettre le pratiquant au coeur de nos préoccupations communes pour mieux coller à la réalité sportive d'aujourd'hui. Je suis convaincue que la politique sportive doit soulever la question du rapport de chacun au sport, afin que chacun, quel que soit son âge, se sente concerné. La politique sportive doit également se mettre au service des autres politiques publiques- santé, qualité de vie au travail, inclusion sociale des personnes handicapées. ensuite considérer le sport comme un bien commun, un bien social qui appartient à tous, État, collectivités, mouvement sportif, monde économique et, bien sûr, pratiquants de tout âge et de toute origine culturelle et sociale. Pour faire vivre cette idée, l'État ne doit plus laisser croire qu'il est le seul promoteur des politiques sportives dans le pays. Il doit devenir un État partenaire du mouvement sportif et des collectivités locales. Pour que le sport se construise en tant que bien commun, il faut arriver à mieux faire ensemble. de démocratiser ce que j'appelle les « primo apprentissages » et donner les clefs aux familles, aux parents, aux grands-parents, aux personnels des crèches, des écoles maternelles et primaires. Il va nous falloir trouver les voies et moyens de parler à tous pour que, dès le plus jeune âge, l'enjeu de la motricité sur le développement de la personnalité soit reconnu à sa juste valeur. Quels outils pour atteindre ces objectifs ? Vous avez tous mentionné la création, au cours du premier trimestre 2019, d'une agence unique chargée, d'une part, de la haute performance et du haut niveau et, d'autre part, du développement des pratiques. Elle remplacera le CNDS et regroupera, pour une prise de décision concertée, tous les acteurs du sport : l'État, le mouvement sportif, les associations de collectivités et le monde économique. Le budget dédié au mouvement sportif et à l'agence est ainsi, pour 2019, évalué à près de 350 millions d'euros, en intégrant les subventions accordées par le ministère des sports au CNOSF et au CPSF. Près de 70 % des moyens d'intervention de cette agence seront dédiés au développement des pratiques. L'enveloppe consacrée à la haute performance sera, quant à elle, en hausse de plus de 40 % par rapport à 2018, avec une enveloppe de crédits portée à 90 millions d'euros J'ai entendu vos inquiétudes quant à l'opérationnalité de l'agence en 2019 et aux potentiels risques de rupture dans le financement des projets sportifs. Je tiens à vous rassurer. à vous rassurer. Sans attendre la nomination prochaine du préfigurateur de l'agence, le ministère des sports travaille déjà actuellement à garantir une continuité de service auprès des acteurs du mouvement sportif. Les opérations pluriannuelles du CNDS, notamment le soutien aux emplois et aux territoires carencés, seront ainsi reprises en totalité par la future agence, tandis que les campagnes de financement au titre de 2019 des projets liés aux parts territoriale et équipements seront relancées, avant même la création officielle de l'agence, afin de continuer à soutenir la pratique sportive dans les territoires. Le budget d'intervention du ministère des sports que je vous présente aujourd'hui sera donc préservé en 2019 par rapport à 2018 et comporte même des mesures nouvelles.

ont pour vocation de conduire des actions nationales et régionales dans le champ du sport et de l'animation. En dehors des personnels pédagogiques et techniques qui continuent à relever de l'État et d'être payés par lui, les agents titulaires des CREPS ont la possibilité d'opter pour une intégration ou pour un détachement dans la fonction publique territoriale d'ici au 1 janvier 2020. Ce détachement sera compensé par l'État aux régions. Entre 2017 et 2020, plus de 10 millions d'euros vont être progressivement intégrés de manière pérenne dans ces dotations générales de fonctionnement versées aux régions.

Vous avez fait voter, madame la ministre, à l'Assemblée nationale, un amendement de 15 millions d'euros en faveur du sport pour tous, notamment pour financer la politique que vous souhaitez mettre en place concernant les piscines et le savoir nager.

en lieu et place des CREPS, elles devraient, par équité de traitement, être accompagnées dans la mise en oeuvre de ces projets. Or tel n'est pas vraiment le cas.

de manière ludique, notamment en raison du matériel spécifique requis, de l'intensité de la pratique, ou des déplacements. Cependant, la France compte 18 millions de licenciés sportifs, pour à peine 15 000 pratiquants inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau.

les crédits entre sport de haut niveau et sport de masse. Loin de moi l'intention

le présente toujours : un modèle en manière de préparation olympique et de double projet, que ce soit pour l'insertion sociale et professionnelle ou pour la recherche du meilleur résultat sportif. Nous ne voterons donc pas cet amendement, qui tend à amputer les crédits affectés au sport de haut niveau.

La trajectoire triennale a donc été ajustée dans le cours de l'examen de ce texte par le Parlement, l'an dernier, afin de tenir compte du besoin de financement supplémentaire né de l'organisation de cette compétition. Cependant, la comparaison entre, d'une part, les crédits supplémentaires inscrits au plafond de dépenses pour les années 2019 et 2020 et, d'autre part, le besoin de financement

de 22 millions d'euros en 2020. Cet écart rompt avec l'engagement du Président de la République. Il menace de surcroît la réalisation des objectifs de développement des pratiques quotidiennes des Français : on attend en effet une progression de 3 millions du nombre de pratiquants d'ici à 2022. Cet écart est d'autant plus préoccupant que les besoins de financement du programme 350 vont considérablement croître lors des prochains exercices. Par rapport à 2019,

20 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement de l'action n° 01, Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques, du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers l'action n° 01, Promotion du sport pour le plus grand nombre, du programme 219 « Sport ». On rétablirait ainsi les crédits destinés au sport pour tous

été volontairement inscrits sur un programme à part afin de garantir l'étanchéité, dont vous rappeliez la nécessité, entre le budget pérenne du ministère des sports et les crédits destinés au financement des équipements. C'est pourquoi les crédits destinés à la SOLIDEO sont en outre budgétés de la manière la plus conforme possible aux prévisions actuelles de programmation. Ils ne pourraient pas être remis en cause par la ponction de 20 millions d'euros que vous proposez, sauf à vouloir compromettre l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

aux taxes affectées. C'est sur ce point, madame la ministre, que vous devez travailler : il faut parvenir à convaincre Bercy de lâcher un petit peu de lest sur ces taxes affectées, parce que le sport doit continuer à être financé par le sport

donc je retire

positionnés sur cet accompagnement scientifique de la performance. C'est l'ANS qui coordonnera à l'avenir l'ensemble des crédits dédiés à la recherche en matière de haute performance. Ce besoin sera donc toujours pris en charge par l'État, mais ce ne sera plus dans le cadre de l'INSEP.

Il apparaît aujourd'hui indispensable d'évaluer l'impact social des politiques sportives et des grands événements sportifs en mesurant leurs coûts et leurs bénéfices réels pour la société. Il ne s'agit pas d'une demande supplémentaire de financement : je souhaite simplement flécher ce type d'études.

son volet intitulé « Le sport conçu comme un investissement social ». Ce type d'études serait particulièrement intéressant pour les organisateurs d'événements sportifs, pour les collectivités territoriales, pour les

Le sujet est extrêmement intéressant, mais la commission a considéré qu'une telle évaluation était déjà possible dans le cadre du programme 219, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la création d'un programme spécifique. Je vous demande donc, mon cher collègue,

déposé cet amendement d'appel. Madame la ministre, il faut clarifier les choses entre la taxe Buffet, la taxe sur les paris sportifs, la « taxe Euro 2016 » qui continue d'être perçue- les recettes arrivent, mais ne sont plus fléchées vers le sport

augmente le plafond de ces taxes. Toutefois, mes années d'étudiant et mes cours de finances publiques m'ont rattrapé : peut-être faut-il rappeler le principe d'universalité budgétaire ? Cet après-midi, on nous disait que les taxes générées par l'eau devaient aller à l'eau ; ce matin que les crédits générés par la transition énergétique devaient aller à la transition énergétique

Son péché originel était d'être distribuée par les parlementaires, ces suppôts de l'ancien monde. On lui a donc coupé la tête sur l'autel de la lutte contre le clientélisme. Comme vous le savez, tous les crédits

titre de la réserve parlementaire. Le FDVA, qui a le mérite d'exister, est précieux pour les rares, très rares, trop rares associations qui en bénéficient. Un décret de juin 2018 en fixe l'organisation. les modalités de répartition sont particulièrement floues et opaques. Les parlementaires n'y ont pas été associés, contrairement à ce qui a été fait pour la DETR. Aujourd'hui, c'est l'autorité préfectorale qui distribue ces fonds. L'objet de cet amendement est simple : il s'agit d'obtenir